La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, avant de vous présenter la position du ministère de l'intérieur sur la proposition de loi, je souhaite profiter de cet instant pour rendre, depuis la tribune du Sénat, un hommage au personnel de la sécurité civile. Son engagement au service des Français est sans faille, quotidien, constant. Un départ en intervention des sapeurs-pompiers a lieu toutes les sept secondes en France. Cet engagement conduit parfois au sacrifice suprême, qui fauche, dans leur jeunesse et dans leur force, des femmes et des hommes engagés au service des autres. heure, je veux commencer par avoir une pensée pour Pierre-François Bonnard, 38 ans, mécanicien opérateur de bord de la base aérienne de Grenoble, mort en intervention il y a dix jours, le 12 septembre. J'ai également une pensée pour Bryan Rimbaut, sapeur-pompier volontaire de 23 ans, décédé en intervention dans la Somme. Ces drames humains illustrent au plus haut point le sens élevé du service public de la grande communauté de la sécurité civile : sapeurs-pompiers militaires, professionnels et volontaires, marins-pompiers, sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile, pilotes et agents du groupement des moyens aériens, fonctionnaires du déminage- chacun, en son grade et qualité, à son poste et à sa responsabilité, au service des Françaises et des Français. Cette tradition de service, cette force de mobilisation, le Gouvernement et les Français les connaissent et les reconnaissent. Je voudrais, avant d'en venir au détail de la proposition de loi, saluer l'action de ces femmes et de ces hommes, qui, tous les jours, portent secours à nos concitoyens. Je crois que, collectivement, nous pouvons en fiers de ce modèle de sécurité civile qui suscite des demandes toujours plus nombreuses de coopération à l'international, fiers d'une organisation solide qui sait toujours s'adapter pour faire face aux nouvelles menaces. Preuve en est la formidable mobilisation de la sécurité civile dans la gestion de la crise sanitaire. Ainsi, quand il a fallu donner un élan nouveau, renforcé, décisif à la campagne de vaccination contre le covid-19, les services d'incendie et de secours ont su se mobiliser selon les directives de la direction générale de la sécurité civile et sous la direction opérationnelle des préfets. Ils sont ainsi présents dans 201 centres de vaccination, dont 119 directement placés sous leur autorité. Aujourd'hui encore, plus de 5 500 sapeurs-pompiers oeuvrent quotidiennement pour vacciner l'ensemble de la population. Lorsqu'il a fallu mettre en place, dans les meilleurs délais, les contrôles aux frontières extérieures pour pratiquer des tests, la force humaine des services d'incendie et de secours et des associations agréées de sécurité civile (AASC) a été, là encore, au rendez-vous. Plus de 820 000 passagers ont été testés par les équipes réparties sur tous les points d'entrée des ports et aéroports internationaux. Cet été, après s'être engagés sur de multiples théâtres extérieurs- Italie, Grèce, Algérie -, nos services d'incendie et de secours, appuyés par les formations militaires de la sécurité civile, sont venus à bout de l'incendie qui ravageait le massif des Maures. Je salue la mobilisation totale des sapeurs-pompiers, leur professionnalisme et leur dévouement exemplaire cet été pour lutter contre les feux de forêt. Cet engagement du quotidien nous oblige. C'est le sens de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers déposée par M. le député Fabien Matras. Cette proposition de loi a été adoptée en mai dernier à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le Sénat en a été saisi dans la foulée et a réalisé un travail de grande qualité. Je veux ici saluer chaleureusement l'investissement sur ce texte des trois rapporteurs : Mme Françoise Dumont, M. Loïc Hervé

Je sais que nous aurons des débats sur certains points, je sais aussi que nous pourrons dégager les consensus utiles. S'agissant de la protection de nos concitoyens, les opinions et les avis divergent peu. En discutant de cette proposition de loi, nous poursuivons tous un objectif commun partagé- largement transpartisan - : offrir le meilleur service de secours aux Français. La proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels apporte- vous le savez parfaitement -des avancées attendues par l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, et que le Gouvernement que le Gouvernement soutient. Consolider notre modèle de sécurité civile, cela signifie avant tout conforter le volontariat et l'engagement citoyen. Le volontariat, c'est cette spécificité française si précieuse qui permet à notre modèle de porter secours à l'ensemble de nos concitoyens, en tout temps, en toutes circonstances et en tous points du territoire. La solidité de ce modèle repose sur les 200 000 femmes et hommes qui, en parallèle de leur travail, de leurs études, de leur vie personnelle ou familiale, volontairement, donnent de leur temps et s'engagent pour secourir les autres. Ces 200 000 femmes et hommes sont, aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels et militaires, le pilier de notre organisation de secours, et ils doivent, je crois, le demeurer. Pour conforter le volontariat, il faut l'encourager et le valoriser. En effet, si l'engagement ne cherche pas la rétribution, il doit être néanmoins reconnu, pour que ce modèle se renforce et perdure. La gratitude de la Nation doit pouvoir s'exprimer pleinement quand les citoyens s'engagent pour la servir et la rendre toujours plus forte et toujours plus unie. Plusieurs mesures figurent dans cette PPL pour aller plus loin dans la reconnaissance et la valorisation du volontariat, l'abaissement du seuil de déclenchement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR). Le ministre de l'intérieur ouvrira d'ailleurs un champ d'échanges avec les financeurs des SDIS pour la revalorisation du montant de la NPFR, qui relève du pouvoir réglementaire. promotion au cadre d'emploi, au grade ou à l'échelon supérieur selon les cas pour les fonctionnaires décédés en service ou grièvement blessés, la création de la qualité de pupille de la République, notamment pour les enfants des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires tués, mise en place de dons de jours de congé au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires. Vous le savez, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin et moi-même sommes d'ardents défenseurs de cet engagement citoyen, qui n'est ni du bénévolat ni du salariat et qui ne doit pas s'en approcher. Il faut à la fois le faciliter, en permettant une meilleure conciliation du volontariat avec l'exercice d'une activité professionnelle, et l'encadrer, pour éviter que certaines pratiques minoritaires ne le déstabilisent. Nous devons aussi et surtout le conforter dans sa spécificité au regard des règles européennes. Après la jurisprudence et à la suite de notre saisine de la Commission européenne, le gouvernement français a obtenu une réponse qui confirme bien la solidité du système du volontariat. La lecture en séance publique au Sénat est l'occasion de mieux prendre en compte dans le texte le rôle essentiel des associations agréées de sécurité civile. C'est pourquoi le Gouvernement soutiendra plusieurs amendements visant, par exemple, à mieux préciser le champ des réserves des services d'incendie et de secours, qui n'ont pas vocation à agir sur le même périmètre de missions que les AASC, ou à réprimer plus efficacement les structures qui, bien que dépourvues d'agréments, se permettent d'agir sur le terrain. Le Gouvernement sera également favorable à l'amendement n°

La meilleure reconnaissance du rôle de ces associations dans cette proposition de loi me semble être une brique majeure apportée par le Sénat. Par ailleurs, cette PPL ne se contente pas de consolider le volontariat. Elle conforte l'ensemble du modèle de sécurité civile, à commencer par les missions des sapeurs-pompiers, qui ont évolué au cours des quinze dernières années en changeant notamment de nature. Le secours d'urgence aux personnes est devenu en quelques décennies l'activité principale des services d'incendie et de secours. Il représente désormais plus de 80 % des interventions. Dans la très grande majorité des cas, les sapeurs-pompiers interviennent en étroite collaboration avec les acteurs de santé, en premier lieu les services du SAMU-centre 15. C'est toujours en totale complémentarité et avec un grand professionnalisme qu'ils interviennent, ensemble, pour offrir le secours le plus rapide et le plus optimal aux victimes. Je tiens à le souligner. souligner. D'une certaine manière, il est urgent de tirer toutes les conséquences de cette évolution en adaptant la loi et nos doctrines opérationnelles aux réalités de terrain. Il y a une certaine urgence à reconnaître les missions des sapeurs-pompiers dans leur globalité, y compris celles qui sont liées aux soins pouvant être prodigués aux personnes secourues. C'est tout le sens de l'article 2 de cette proposition de loi. La proposition de loi traite également dans son article 3 du sujet majeur des carences ambulancières, enjeu important du fonctionnement actuel des services d'incendie et de secours. L'Assemblée nationale a aussi permis aux SIS de retrouver la maîtrise et la hiérarchisation de leurs moyens en permettant la temporisation de l'engagement. La commission des lois du Sénat a souhaité introduire la requalification. Sur ce dernier point, il semble important au Gouvernement de respecter les équilibres trouvés entre les services d'incendie et de secours et les structures d'aide médicale d'urgence. C'est pourquoi le Gouvernement proposera un amendement de rétablissement du texte de La proposition de loi apporte aussi beaucoup en matière de doctrine d'intervention, d'organisation et de fonctionnement des services d'incendie et de secours. Ainsi, le Gouvernement a porté des amendements sur les pactes capacitaires et les contrats territoriaux de réponses aux risques et aux effets de menaces à l'Assemblée nationale. Nous soutiendrons devant le Sénat des amendements visant à élargir les communes soumises à la réalisation obligatoire d'un plan communal de sauvegarde. Les expériences récentes nous montrent à quel point un PCS, même simple, et des exercices réguliers peuvent réussir à sauver des vies. Car c'est bien de cela qu'il s'agit ! C'est cela qui doit guider nos réflexions et notre action.

L'article 9 de la proposition de loi traite de la modernisation de notre dispositif de prévention. Le déploiement du, que nous avions annoncé pour 2022, viendra améliorer en temps réel l'alerte et l'information des populations en cas de survenance d'un événement majeur. Il permettra une diffusion massive, prioritaire et rapide aux populations exposées à un risque des informations essentielles à leur protection. Cette proposition de loi est ainsi devenue au gré des apports successifs- de l'Assemblée nationale hier, du Sénat aujourd'hui et dans les prochains jours, et et du Gouvernement constamment -le support juridique d'une rénovation profonde de notre modèle de sécurité civile dans un objectif toujours partagé d'excellence opérationnelle

Nous aurons de riches et féconds débats avant d'y parvenir, mais je ne doute pas que nous parviendrons ensemble à atteindre l'objectif attendu. La parole

depuis de nombreuses années, la commission des lois donne à la sécurité civile la place primordiale qu'elle mérite. C'est la raison pour laquelle elle a désigné, pour cette proposition de loi, trois rapporteurs appartenant aux trois principales sensibilités politiques de notre assemblée. Cette configuration aurait sans doute été impossible sur d'autres sujets, ou en d'autres lieux, mais elle n'a posé aucun problème, donné lieu à aucune dissension, tant nous savons à quel point les enjeux de cette proposition de loi sont fondamentaux pour notre nation tout entière. Je tiens ici à remercier chaleureusement Loïc Hervé et Patrick Kanner, grâce à qui la qualité de notre travail a été, je pense, à la hauteur des enjeux. enjeux. Initialement déposé par le député Fabien Matras, puis soutenu par le Gouvernement, ce texte entend se placer dans la lignée des grandes lois de sécurité civile, au même titre que la loi de 1996 relative aux services d'incendie et de secours ou celle de 2004 portant modernisation de la sécurité civile. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à considérer que certaines dispositions du texte transmis par l'Assemblée nationale étaient de véritables avancées qu'il ne fallait pas remettre en cause par pur principe. Cette objectivité nous conduit à partager un certain nombre de points de vue avec le Gouvernement. En revanche, nous avons été particulièrement vigilants lors de l'examen des dispositions qui n'emportaient pas de consensus à leur sortie de l'Assemblée nationale. Les plus sensibles concernent l'expérimentation des plateformes communes de réception des appels d'urgence. L'article 31 de la proposition de loi initiale prévoyait la mise en place du 112 comme numéro d'appel d'urgence unique ainsi que la mutualisation des plateformes de réception des appels d'urgence. Très attendu par les acteurs de la sécurité civile, ce dispositif a toutefois soulevé de vives protestations de la part des acteurs de la santé, qui y ont vu une remise en cause possible du principe de la régulation médicale et du service d'accès aux soins récemment mis en place. La commission des lois ne remet pas ici en question son souhait de voir aboutir, à terme, un numéro unique et des plateformes communes. Ce souhait a d'ailleurs été conforté par notre déplacement sur la plateforme commune de réception des appels d'Annecy. Toutefois, nous avons considéré que les conditions n'étaient, pour l'heure, pas réunies pour la mise en place définitive d'un tel système sur l'ensemble du territoire national. La commission a donc conservé le principe d'une expérimentation, mais a apporté des modifications, dont certaines sont à nos yeux clairement indispensables. La première concerne la prise en compte des associations agréées de sécurité civile dans le dispositif dont elles étaient exclues, et ce malgré le caractère incontournable de leurs actions. La deuxième tend à mettre les présidents des SDIS concernés sur le même plan que le représentant de l'État ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans la mise en oeuvre et l'évaluation des expérimentations. Enfin, la troisième tend à prévoir qu'en cas de succès de l'expérimentation un référentiel national relatif au fonctionnement des plateformes serait élaboré par l'ensemble des acteurs concernés, dans le respect des prérogatives de chacun. Cette logique de dialogue et d'échange semble impérative pour mener à bien un tel projet de mutualisation. Madame la ministre, ces modifications ne relèvent que du seul bon sens. Pourtant, vous souhaitez toutes les remettre en cause, sans exception, par un amendement que vous avez déposé. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard.

La posture- permettez-moi cette expression -du Gouvernement quant aux avancées de la commission des lois m'interpelle. De notre côté, nous avons su saluer les avancées du texte transmis au Sénat. Je fais ici référence aux articles 1, 2 et 3, qui clarifient utilement le cadre d'intervention des services d'incendie et de secours- sous certaines réserves, comme l'expliquera Loïc Hervé. Je fais également référence aux articles 20 et 21 : le premier prévoit des promotions à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels décédés lors de leur service ou ayant réalisé des actes de bravoure ; le second crée une mention « Mort pour le service de la République » au bénéfice de personnes appartenant à des corps ou entités habituellement exposés à des situations de danger, tout en ouvrant le nouveau statut de « pupille de la République » pour leurs orphelins. leurs orphelins. Malgré vos salutations amicales, madame la ministre, nous ne sommes pas naïfs. Le projet de loi déguisé que nous examinons aujourd'hui a mis près d'un an à être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Son examen a été reporté de mois en mois, car le Gouvernement n'y trouvait pas, à l'époque, d'intérêt immédiat. d'intérêt immédiat. Si la procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement, si ce texte qui concerne directement les départements a été transmis au Sénat en plein milieu des élections départementales, si nous avons dû l'examiner en commission au mois de juillet, au pas de course, sous une grêle de projets de loi, et si une CMP va être convoquée dans des délais record, c'est seulement parce que le congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers se tiendra au mois d'octobre à Marseille

Nos attentes vis-à-vis du Gouvernement dépassent ce texte. Je fais ici référence à la jurisprudence- évoquée par notre collègue Françoise Dumont et par vous, madame la ministre -qu'il n'est plus besoin de présenter dans notre hémicycle et par laquelle la Cour de justice de l'Union européenne considère que les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être assimilés à des travailleurs. Certes, l'article 22 A de la proposition de loi tend à contrer cette jurisprudence- vous l'avez rappelé -, mais son niveau législatif le rend parfaitement inopérant face à une jurisprudence de niveau européen. Ce texte est l'occasion pour nous de demander au Gouvernement s'il compte soumettre une réponse juridique effective à ses partenaires européens, à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. C'est l'occasion ou jamais de faire bouger les lignes. Madame la ministre, vous l'aurez compris, nous sommes là pour défendre l'intérêt général. Vous pouvez compter sur nous. Or l'intérêt général ne se résume pas à la course contre la montre que vous nous imposez dans le cadre de l'agenda parlementaire. Sachez néanmoins que nous serons constructifs afin de préserver la sécurité civile de notre pays. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, l'arrêt et l'expérimentation des plateformes uniques n'ont pas été les seuls sujets d'attention de la commission des lois.

les SDIS réalisent des transports sanitaires pour pallier l'absence d'autres moyens, dont ceux des ambulanciers privés. Ces carences sont dénoncées par les acteurs de la sécurité civile, car, d'une part, la qualification d'une mission en carence relève principalement de de l'appréciation du médecin régulateur du SAMU et, d'autre part, le montant de l'indemnisation des SDIS s'élève à 123 euros par carence alors que le coût moyen qu'ils supportent est estimé entre 450 et 500 euros. En outre, ces créances sont parfois difficilement recouvrées par les SDIS., le développement de ces carences ajouté à leur mauvais remboursement conduit à un transfert de charges de fait entre le niveau national, qui finance les SAMU, et les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les départements et les communes, qui financent les SDIS. Nous avons donc été très favorables à l'article 3 de la proposition de loi, qui donne une définition objective de la carence ambulancière. C'est une vraie avancée qu'il faut reconnaître. Néanmoins, la commission des lois a jugé utile d'adopter un amendement qui tend, d'une part, à supprimer l'obligation de prescription médicale pour pouvoir qualifier une intervention de carence ambulancière et, d'autre part, à rétablir la possibilité de procéder à la requalification de cette carence. Cette précision permettra aux SDIS d'être justement indemnisés lorsqu'ils ont réalisé une intervention à la demande du 15 dont il s'est avéré, par la suite, qu'elle relevait en pratique de la carence ambulancière.

Enfin, je souhaite finir sur des points positifs, puisque certains apports de la commission des lois n'ont pas fait l'objet d'amendements ni du Gouvernement ni de votre part, mes chers collègues. Le premier porte sur la mise en place de référents « sécurité » au sein des SDIS. Ils seront notamment compétents pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs-pompiers. Il s'agit de l'une des propositions du rapport de la commission des lois de 2019 sur la sécurité des sapeurs-pompiers. Le second concerne la possibilité ouverte à l'ensemble des conseillers municipaux de représenter leur commune ou leur EPCI au conseil d'administration du SDIS, faculté ouverte actuellement uniquement aux maires ou à leurs adjoints. Cet apport fait écho à la création, par la proposition de loi, d'un correspondant « incendie et secours » au sein de chaque conseil municipal. Madame la chers collègues, ce dernier point me pousse à être optimiste quant à l'avenir de ce texte. Nous sommes convaincus que la sagesse du Sénat ne manquera pas de persuader nos collègues députés. C'est, en tout cas, le souhait que nous formulons, avec Françoise Dumont et Patrick Kanner.

les attentes face à ce texte sont immenses et nombreuses, non seulement pour les acteurs du secteur, mais aussi pour notre modèle de sécurité civile et son bon fonctionnement. Les débats à l'Assemblée nationale

de préserver et de valoriser notre système de secours et de sécurité civile. Le meilleur moyen d'y parvenir est de travailler à son amélioration et d'en assumer une réforme. Le contexte dans lequel nous vivons est malheureusement marqué par une hausse importante des violences envers les sapeurs-pompiers, dont le sentiment d'insécurité durant les interventions ne cesse de croître. Je rappelle des chiffres déjà bien connus : entre 2017 et 2018, l'augmentation agressions a été évaluée autour de 25 %. Cela n'est pas acceptable au sein de notre société, d'autant que les sollicitations augmentent elles aussi et sont parfois assez éloignées des domaines d'activité premiers des sapeurs-pompiers. Le texte que nous examinons paraît revêtir un équilibre intéressant. Les articles relatifs à la question des retraites, de la réserve citoyenne ou encore aux autorisations d'absence pendant le temps de travail vont dans le bon sens. Je souhaite évoquer plusieurs points qui me semblent essentiels, par rappeler le rôle des sapeurs-pompiers volontaires, acteurs ô combien indispensables en milieu rural. Leur recrutement doit être facilité à la fois dans le secteur public et au sein des entreprises. Plusieurs articles sont consacrés à leur place en entreprise : c'est un bon moyen de valorisation. l'aménagement du temps de travail et la flexibilité des jours de repos non pris afin de permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'assurer leurs missions et activités sont des avancées intéressantes. Je proposerai des amendements d'amélioration allant dans le même sens.

que la gestion des appels et les décisions prises en matière de santé restent entre les mains du seul médecin régulateur du SAMU. Enfin, je ne peux pas clore mon propos sans évoquer un sujet essentiel pour notre modèle de sécurité civile, civile, particulièrement pour les sapeurs-pompiers volontaires : le fait de ne pas assimiler leurs activités à celle d'un travailleur. C'est l'un des objectifs de l'article 22 A de cette proposition de loi. Nous comprenons que la portée juridique limitée de cet article ne résoudra pas le problème provoqué par la jurisprudence européenne et la directive relative à la durée du temps de travail. Concernant l'activité des sapeurs-pompiers volontaires, j'ai moi-même posé la question à plusieurs reprises au Gouvernement durant les deux dernières années. La réponse de la Commission européenne au ministre de l'intérieur, bien que donnant des éléments de réponse concrets, n'est pas satisfaisante, car elle n'exonère pas totalement les sapeurs-pompiers volontaires, elle propose seulement une interprétation au cas par cas. Comme le définit la loi du 20 juillet 2011, « l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel Et c'est ce que souhaitent les sapeurs-pompiers volontaires et toutes les collectivités territoriales rurales ! Madame la ministre, il y va de la pérennité des centres de secours en milieu rural. La présidence française du Conseil de l'Union européenne doit absolument apporter des solutions concrètes Ce texte doit apporter des avancées significatives pour les sapeurs-pompiers et pour le modèle que la France peut s'enorgueillir de développer. La proposition de loi a été enrichie, notamment par son passage en commission,

Notre modèle de sécurité civile connaît des difficultés et a besoin de réponses concrètes. Plusieurs constats ont été pris en compte dans notre réflexion. Le premier concerne le volontariat : l'engagement volontaire, vital dans notre système, est trop peu reconnu et parfois mis en difficulté, comme nous avons pu le constater à l'occasion d'une décision européenne récente. La présente proposition de loi a le mérite de chercher à redéfinir et à consolider le rôle et le champ d'action des pompiers.

Personne ne peut le nier, le nombre d'épisodes extrêmes est en hausse : pluies violentes, incendies, épisodes de chaleur, autant de situations qui exigent la participation de nos services départementaux d'incendie et de secours J'en profite pour remercier ici ces héros du quotidien qui, trop souvent au péril de leur vie, viennent en aide à la population et combattent les feux qui ravagent de plus en plus nos territoires ou ceux de nos voisins européens, réduisant parfois à néant des années d'efforts de protection de la biodiversité. En outre, la récente crise du covid a montré une forte mobilisation des pompiers dans les transports sanitaires comme dans l'appui, voire dans l'organisation de la campagne de vaccination. En dehors de cette crise inédite, la situation sociale et sanitaire de notre pays a évolué ces dernières années. Les pompiers sont souvent le dernier recours face à une détresse qui reflète de trop nombreuses inégalités, particulièrement face à l'accès aux soins. Le texte présenté aujourd'hui donne les outils nécessaires aux SDIS pour mieux travailler en coordination avec les SAMU dans le cadre des soins de secours aux personnes. Toutefois, les articles qui s'y attachent, s'ils constituent une avancée, ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Alors que certains évoquent et recherchent un renforcement de la chaîne pénale, peu se penchent sur la chaîne sanitaire. Les débats en commission ont mis en avant les difficultés liées aux carences ambulancières. Quel que soit l'opérateur chargé de ce transport sanitaire, l'entonnoir se déverse toujours sur les urgences hospitalières publiques. L'hôpital était déjà à bout de souffle avant même les deux dernières années, qui ont été encore plus difficiles. Si ce texte touche du doigt le sujet de ces transports, on n'y trouve aucune réflexion sur les possibilités de développer les services d'accès aux soins. Certes, un article permet l'expérimentation de plateformes communes de réception d'appels d'urgence

Au-delà de ces réflexions sur la philosophie générale du texte, permettez-moi d'évoquer quelques questions qui restent en suspens. S'agissant de la coordination avec les maires et les préfets, les acteurs locaux doivent avoir droit à la parole sur l'organisation. La mobilisation transpartisane ayant permis, par exemple, le maintien des canadairs sur la base de Marignane en est un exemple. Notre groupe proposera plusieurs amendements à ce sujet, dont certains concernent Marseille, qui, comme Paris, bénéficie d'une protection par les militaires que sont les marins-pompiers.

Le groupe Écologiste- Solidarité et Territoires souhaite une valorisation accrue du volontariat et proposera que cela passe aussi par une bonification lors des examens dans l'enseignement pour les volontaires mineurs faisant preuve d'une implication citoyenne forte. Enfin, afin de reconnaître à leur juste valeur les sacrifices de certains, nous proposerons une modification visant à élargir les circonstances conduisant à la reconnaissance du statut de pupille de la République pour les orphelins de ces acteurs morts dans le cadre de leur service.

malgré quelques réserves et en formant le voeu que ses apports soient intégrés, le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires votera ce texte.

le déploiement de la stratégie vaccinale, sans oublier les innombrables interventions de proximité et de secours à la personne : ces proches réalités sanitaires et climatiques illustrent le rôle essentiel et la diversité des interventions de la sécurité civile dans nos territoires.

mais aussi celui de tous les sapeurs-pompiers décédés en mission. Le dénominateur commun de cette pluralité est en effet l'engagement, socle de notre modèle de sécurité civile, dans lequel les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou, pour près de 80 % d'entre eux, volontaires, occupent une place essentielle. ce modèle, les 250 000 femmes et hommes pompiers donnent en gage leur personne pour la prévention des dangers, mais aussi pour l'aide et le secours à leurs concitoyens en péril, un engagement républicain qui porte haut le principe de fraternité et, plus encore, le donne à voir dans sa réalisation concrète et quotidienne. Ce modèle fait face, aussi, à de nombreux enjeux que prend en compte la proposition de loi de notre collègue député Fabien Matras, que nous examinons aujourd'hui, dix-sept ans après la dernière grande loi de modernisation de la sécurité civile. civile. Parmi ces enjeux, relevons la diversité croissante des missions des sapeurs-pompiers, marquées, notamment, par l'augmentation des interventions au titre du secours à la personne ou la dégradation de leurs conditions d'opération en raison de la hausse des violences dont ils font l'objet, qu'avaient utilement soulignée nos rapporteurs Loïc Hervé et Patrick Kanner dans un précédent rapport. à l'esprit la crainte qu'a suscitée, en 2018, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne s'agissant de la conception du statut de sapeur-pompier volontaire, indissociable de notre modèle de sécurité civile. Mme la ministre a utilement apporté certaines clarifications devant l'Assemblée nationale et, à l'instant, dans notre hémicycle ; le débat, complexe, se poursuivra lors de l'examen de nombreux amendements. Mes chers collègues, je ne serai pas exhaustif à propos des presque soixante-dix dispositions comprises dans la proposition de loi, dont la majorité- il faut le souligner -fait l'objet d'une convergence de vue entre les deux assemblées et les différents groupes politiques qui les composent. Ce texte permet tout d'abord de reconnaître et d'intégrer dans la loi la réalité opérationnelle des interventions des sapeurs-pompiers, en faisant figurer parmi les missions des services d'incendie et de secours les soins d'urgence. Il permet ensuite de consolider le volontariat en valorisant et en reconnaissant cet engagement à sa juste valeur. Je pense notamment, sur le plan social, à l'extension de l'accès à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance,

La juste reconnaissance de l'engagement des sapeurs-pompiers passe également par les garanties de leur protection physique, que le présent texte, tel qu'il nous est arrivé de l'Assemblée nationale, propose de renforcer en étendant la constitution de partie civile par les SDIS et la possibilité d'indemnisation à tous les cas d'incendies volontaires, en durcissant les peines encourues pour outrage à un sapeur-pompier dans l'exercice de sa mission ou, encore, en généralisant l'usage des caméras individuelles et en instaurant dans chaque SDIS un référent « sécurité Ces dispositions s'ajoutent à la limitation, prévue dans un autre véhicule législatif, des réductions de peine accordées en cas d'infraction commise sur un sapeur-pompier. Texte de reconnaissance, cette proposition de loi est aussi un texte d'équilibre, cohérent

participent au lien social, mais sont également confrontés au défi des vocations et de l'engagement. De même, la définition positive des carences ambulancières permettra de clarifier le régime des interventions ne relevant pas de la compétence des SDIS, afin que les dépenses ne se rattachant pas à l'exercice de leurs missions ne pèsent pas sur les collectivités territoriales. Cet enjeu sera également traité au niveau des conventions entre SDIS et SAMU, maillons indispensables et complémentaires de la chaîne du secours. En effet, cette proposition de loi ne peut pas tout régler, et les conditions de sa mise en oeuvre seront décisives. Cette remarque s'applique également au déploiement de la télétransmission des constantes médicales depuis les véhicules dans le cadre des interventions de secours, prévu dans le texte. Enfin, soulignons la mise en oeuvre d'une plateforme commune de traitement des appels et l'expérimentation de plusieurs configurations de regroupement de numéros d'urgence. Il s'agit, sans supprimer la nécessaire régulation médicale, d'aboutir à une solution garante d'une plus grande lisibilité et d'une meilleure efficacité dans la prise en charge des situations d'urgence. Cela implique de recourir à une expérimentation, dont les modalités pourront encore faire l'objet de débat, mais dont le principe nous réunit. C'est C'est dans un même souci de protection et d'efficacité que nous soutiendrons les amendements portés par le Gouvernement visant à renforcer l'obligation d'acheminement des communications d'urgence, dans la continuité des préconisations de l'Anssi à la suite de la grave panne intervenue au mois de juin dernier. Mes chers collègues, plusieurs débats entamés en commission se poursuivront dans notre hémicycle ce soir, mais je veux saluer l'esprit de consensus qui a présidé à l'élaboration et à l'examen de cette proposition de loi, comme en témoignent les 500 cosignatures dont celle-ci a fait l'objet à l'Assemblée nationale, et m'y associer. Le groupe RDPI la soutiendra donc en espérant vivement

nous arrivons au terme d'un été au cours duquel nos sapeurs-pompiers auront, hélas ! été sollicités sur de nombreux fronts. Je pense notamment à ceux qui ont lutté contre le feu qui a dévasté près de la moitié de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures. Aussi, je voudrais dire avant tout mon admiration et ma reconnaissance pour ceux qui forment ce corps. Face à leur engagement, il était impératif que le législateur réponde avec force pour dire combien nous sommes déterminés à les soutenir. De ce point de vue, j'ai le sentiment que cette proposition de loi est à la hauteur des objectifs. Les premiers apports du Sénat, à travers les travaux de notre commission des lois, ont permis de lui donner la densité attendue par ceux qui offrent une partie de leur vie et de leur temps à notre nation. Parmi les mesures qui ont pu faire l'objet d'une attention particulière chez les membres du groupe du RDSE, j'ai en particulier à l'esprit l'article 31 et l'expérimentation de la mise en place de plateformes communes de réception des appels et d'un numéro unique d'urgence. Les représentants des sapeurs-pompiers ont souligné combien ce dispositif non seulement serait utile à leur service, mais répondrait plus largement à un besoin collectif de notre société. Certes, nous avons le sentiment que le texte aurait pu être encore plus complet en prévoyant directement, comme c'était initialement le cas, que le numéro unique en question serait le 112. Il demeure que le dispositif prévu doit être salué. Il faut également souligner l'article 30, portant la création du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers », attribué aux employeurs publics ou privés ayant conclu une convention de disponibilité. Le texte, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, manquait peut-être d'ambition aussi, je me réjouis des apports de notre commission instituant un dispositif bien plus abouti à travers l'exonération de charges patronales pour les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Ce mécanisme est attendu par l'ensemble des acteurs, afin de faciliter concrètement les conditions d'engagement. Nous espérons donc qu'il puisse être maintenu jusqu'au terme de la navette parlementaire. voudrais désormais aborder un point spécifique : la question de l'engagement de notre jeunesse et de sa sensibilité aux questions de sécurité civile. Les moyens mis en place pour l'encourager nous semblent encore insuffisants et risquent, à terme, de provoquer un essoufflement des effectifs. Il nous semble, par exemple, en vue de promouvoir la vocation de sapeur-pompier auprès des jeunes et de réussir leur formation, qu'il faudrait développer davantage les sections études de jeunes sapeurs-pompiers volontaires. ceux qui n'envisageraient pas un parcours scolaire aussi spécifique, il paraît impératif que tous les élèves bénéficient d'une sensibilisation à l'engagement de sapeur-pompier volontaire. D'une autre façon, lorsque nos jeunes ont fait le choix d'être volontaires, la valorisation de leur service pourrait passer par la validation des acquis de l'expérience. Bref, à travers ces illustrations, la question de la jeunesse ne devra pas nous échapper, et je nourris l'espoir que nos débats permettent d'avancer encore. encore. Si cette proposition de loi était adoptée, cela ne permettrait toutefois pas de régler l'ensemble des difficultés auxquelles font face nos services. Les échanges que j'ai pu avoir avec différents acteurs de terrain m'ont permis de faire certains constats. La culture des premiers secours et des premiers gestes se perd progressivement et traduit une forme d'échec des pouvoirs publics, qui ne parviennent pas à les transmettre à l'ensemble de nos concitoyens. Cela se manifeste très concrètement sur nos territoires lorsque certains de nos concitoyens ne savent pas comment réagir face à une catastrophe telle qu'un incendie ou une inondation. De la même façon, la sursollicitation des pompiers, au détriment des cabinets médicaux, lorsqu'il n'y a pas de véritable urgence est un échec de notre société, qui a perdu la culture de ses services de secours et d'urgence et ne parvient plus à savoir quand les appeler sans excès.

de rendre un hommage consensuel à ces hommes et à ces femmes qui assurent la sécurité civile de notre quotidien ; je m'incline ici devant la mémoire de celles et ceux qui ont perdu leur vie dans l'accomplissement de leur mission. qu'on ne peut pas omettre ce soir de souligner que la dernière loi de gestion de la crise sanitaire a quelque peu abîmé le lien de confiance entre l'État et nos soldats du feu. Le fonctionnement de notre modèle de sécurité civile évolue, la crise y a, pour partie, contribué. Dès 1789, la Garde nationale révolutionnaire a cultivé les valeurs du volontariat cet engagement citoyen, attaché au statut de pompier volontaire, est aujourd'hui en crise depuis une dizaine d'années. Les effectifs de volontaires continuent de stagner ou de diminuer, et nous attendons le bilan du Gouvernement après les trente-sept mesures de revalorisation La directive européenne de 2003 sur le temps de travail et la jurisprudence de 2018 menacent ce pilier de notre sécurité civile, mais révèlent aussi les limites actuelles et les besoins de revalorisation du statut de volontaire. Le sous-effectif chronique des pompiers professionnels conduit à utiliser de manière abusive le statut de volontaire afin de contourner les droits sociaux concernant le temps de repos ou le paiement des indemnités. Pour reprendre le témoignage d'un pompier relevé par le sociologue Romain Pudal, « le SDIS est un qui vit de la précarité des volontaires ». Ces volontaires représentent 79 % de nos pompiers et assurent une action de proximité primordiale. Nous souhaitons faire perdurer cet engagement citoyen, mais sans que celui-ci devienne pour autant un substitut aux pompiers professionnels pour des raisons de restrictions budgétaires. Le double statut professionnel et volontaire manque d'encadrement et permet des cumuls d'heures qui créent de l'insécurité lors des interventions, mettant directement en danger la santé de nos pompiers. Pour que notre modèle de sécurité civile perdure, la revalorisation du volontariat doit passer par un meilleur traitement des volontaires, sans lequel les vocations peineront à se renouveler. La présente loi y contribue par certaines revalorisations et certaines protections ainsi que par une meilleure reconnaissance. Toutefois, sans professionnalisation, rien ne se fera, car nous retomberons toujours sur ce problème structurel d'effectifs de professionnels Une réflexion plus poussée sur les moyens mis en oeuvre est donc nécessaire. Reconsidérer les statuts, c'est aussi prendre en compte l'évolution des missions des pompiers. Le secours à la personne est aujourd'hui leur première activité et concerne 85 % des missions. Cela implique d'en redéfinir le périmètre, notamment vis-à-vis d'autres services, comme l'aide médicale d'urgence, point sur lequel la proposition de loi comporte plusieurs avancées. Le changement de nature de ces missions met les pompiers face à de nouveaux risques et implique un nouveau rapport entre pompiers et population. Nous déplorons l'explosion des agressions envers les pompiers et nous estimons que leur faire porter des caméras ne réglera en rien les causes premières de ce phénomène. Valoriser le métier de pompier, c'est aussi, selon nous, mieux les former et mieux distinguer leurs missions de celles des forces de l'ordre afin de mieux les protéger en amont. La vraie lacune de cette proposition de loi est l'absence de dispositions financières. Les budgets des SDIS sont fortement corsetés, la crise ne fait que peser davantage sur les finances locales, alors que les ressources humaines et financières manquent. Depuis 2000, le nombre de centres d'incendie et de secours chute, compromettant l'égal accès sur l'ensemble du territoire aux interventions et aux soins urgents. Nous sommes passés de 8 700 centres en 2002 à 6 227 centres aujourd'hui ; cette perte de proximité freine l'engagement de pompiers volontaires. À cette mise en danger de nos concitoyens s'ajoutent des problèmes de sécurité liés à la baisse des dépenses d'investissement dans le matériel. L'État doit être le correcteur de ces inégalités et de ces dangers, mais, depuis 2017, on constate une chute de 60 % de la dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours. Le Gouvernement se permet même d'afficher politiquement la revalorisation de la prime du feu, financée en réalité par les départements, qui sont à bout de souffle. Nous voterons ce texte, qui permet plusieurs petites avancées et apporte des précisions bienvenues. L'examen des articles nous donnera l'occasion de nous exprimer sur l'ensemble de ces dispositions, dont certaines nous posent question, notamment en l'absence d'étude d'impact.

Vérien. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, que serions-nous dans nos campagnes sans nos sapeurs-pompiers volontaires ? Comment pourrions-nous être correctement protégés sans nos centres de secours, bien sûr, mais aussi sans nos CPI au maillage territorial extrêmement fin ? fin ? S'il fallait salarier tous nos pompiers, aurions-nous encore une équipe d'une dizaine de sapeurs, hommes et femmes, dans un village de 330 habitants, comme Sainpuits, dans l'Yonne sont pas là que pour la Sainte-Barbe, ce sont des pompiers opérationnels, qui sauvent des vies, souvent, et des granges, parfois. Nos pompiers, nous en avons besoin. C'est simple : leurs interventions sont en constante augmentation, avec 26 % de sollicitations opérationnelles en plus entre 2011 et 2017.

et l'efficacité de notre sécurité civile et laisserait nos villages dans le désarroi. C'est pourquoi ce texte est utile, qui entend revaloriser l'engagement des pompiers, lequel va parfois jusqu'au don de leur vie. En dix ans, 102 pompiers sont morts en service, et il est primordial que la Nation leur témoigne toute la reconnaissance qui leur est due. Les promotions à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers décédés lors de leur service comme le sont le nouveau statut de pupille de la République pour leurs orphelins et la clarification de la notion d'accident de service, pour une meilleure prise en charge des volontaires par la sécurité sociale. Sachez que les pompiers eux-mêmes savent se prendre en main ; je parlais de l'Yonne, dans le centre de secours de Saint-Sauveur-en-Puisaye, l'une des pompiers organise tous les ans une soirée Zumba au bénéfice des orphelins des pompiers. L'autre difficulté, après le recrutement de pompiers volontaires, est de trouver des entreprises partenaires. C'est pourquoi les mesures permettant de faciliter l'attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » ainsi que les réductions d'impôt et de cotisations sociales qui y sont attachées sont les bienvenues. Les communes jouent souvent le jeu, mais il est vrai que, lorsqu'un pompier sort

qu'elle ne permet pas de traiter le problème structurel d'une présence trop faible des services de soins et qu'elle détourne les pompiers de leur véritable rôle, cette mission est très mal indemnisée, bien en deçà du coût réel supporté par les SDIS.

Ce texte ne vise pas seulement à corriger des phénomènes qui nuisent au développement de notre modèle de sécurité civile, il entend également faire évoluer ce modèle et le moderniser. Ainsi, il fait écho au souhait d'une plus grande diversité des profils, à travers, par exemple, un objectif de parité au sein des conseils d'administration du SDIS. Aujourd'hui, les femmes ne représentent que 10 % des effectifs des sapeurs-pompiers ; on peut faire mieux, pour preuve Saint-Sauveur-en-Puisaye, 930 habitants, un centre de secours, une trentaine de pompiers, tous volontaires, dont douze femmes. Non, un pompier, ce n'est pas seulement un Superman qui sait vaincre le feu, c'est aussi une femme ou un homme qui assiste une personne en détresse, une femme qui accouche ou un enfant blessé ! Cette pluralité sociale et sexuée permet de faire face à des situations plus diverses. Il est également prévu une revalorisation de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. L'amélioration matérielle de l'engagement de nos sapeurs-pompiers constitue toujours une avancée. Je voudrais malgré tout aborder le sujet de l'allocation de vétérance. Dans le cas des pompiers communaux, cette allocation est entièrement payée par la commune. Si elle vient légitimement récompenser des années d'engagement, elle pèse lourdement sur les finances de certains villages, alors qu'ils ont pourtant à coeur de maintenir un service de secours et d'incendie au plus proche du territoire et des citoyens. Cette philosophie est d'ailleurs partagée par les pompiers, souvent très attachés à leur commune, et qui ne souhaitent pas forcément rejoindre le corps départemental. Communes rurales et pompiers ne devraient donc pas avoir à choisir entre le maintien d'un service de secours de proximité et la juste récompense d'années d'engagement au service des autres. Cette situation est d'autant plus regrettable que les prestations versées pour les pompiers rattachés au corps départemental sont financées, elles, pour moitié par l'État. En outre, il est impossible pour le SDIS de prendre en charge tout ou partie du financement de l'allocation de vétérance pour soulager les communes, car c'est illégal. Il serait donc utile de donner aux départements la possibilité de soutenir les communes dans le financement des allocations de solidarité. Malheureusement, l'article 40 est là, qui veille et retient des amendements pourtant attendus par de nombreuses communes rurales, ce qui fait que les seuls que vous verrez seront des demandes de rapport, mais, bien entendu, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Autre sujet très sensible dans mon beau département de l'Yonne : la plateforme commune d'appel 15-18, souhaitée tant par les « rouges » que par les « blancs », mais qui nous est pour l'instant refusée par l'ARS, préférerait supprimer le 15 départemental pour le transférer à la région, comme elle l'a déjà fait pour la Nièvre. Je suis donc particulièrement satisfaite de voir dans cette proposition de loi l'expérimentation d'un numéro unique qui regrouperait, selon les configurations, pompiers, policiers et SAMU, ou seulement pompiers et SAMU. Faut-il regrouper le 15, le 17 et le 18, ou seulement le 15 et le 18 ? Là encore, cette proposition pragmatique envisage différentes configurations, ce qui permet à chacun d'aller au plus loin, en fonction de ses spécificités locales. En tout cas, je le répète, au nom de toutes les forces vives de l'Yonne, que ce soit les élus, les médecins, les pompiers, nous sommes prêts pour un 112 Vous l'aurez compris, je suis admirative de nos pompiers, plus particulièrement de nos pompiers volontaires. Ils sont une force et un besoin pour nos territoires. Ils ont aujourd'hui besoin de nous pour améliorer leur situation. En conséquence, même s'il reste des points de vigilance, le groupe Union Centriste votera ce texte.

Var, plus de 1 000 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Dans le territoire dont je suis l'élu, cinq sapeurs-pompiers ont prêté main-forte. Oui, la sécurité civile appelle une contribution de tous ! Elle appelle aussi un consensus politique, au-delà de la diversité de notre assemblée. Nous joindrons notre voix à toutes celles qui rendent hommage aux soldats du feu. Nous regrettons seulement que ce texte arrive si tard dans le calendrier législatif. Des esprits plus malicieux que le mien estimeront sans doute qu'il intervient au contraire juste au bon moment. Cependant, nous ne mégoterons pas notre soutien à cette proposition de loi, qui poursuit un objectif clair : consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Ce texte présente, à mon avis, deux séries d'avancées notoires : d'une part, reconnaître et, d'autre part, pérenniser l'engagement des sapeurs-pompiers. Reconnaître l'engagement des sapeurs-pompiers, c'est d'abord reconnaître leur pleine capacité d'action dans le cadre de leurs interventions. La proposition de loi dit enfin ce que sont les opérations de secours et reconnaît aussi la capacité des sapeurs-pompiers à prodiguer certains soins d'urgence. Reconnaître l'engagement des sapeurs-pompiers, c'est rendent à notre République. L'engagement des sapeurs-pompiers est un engagement périlleux. Leur exposition accrue face au développement des événements climatiques extrêmes appelle une reconnaissance du service rendu. parce qu'elle est symbolique, doit aussi être forte. La proposition de loi porte la création de la mention « Mort pour le service de la République ». Cette reconnaissance doit également être effective. La proposition de loi porte aussi la création du statut de « pupille de la République » pour les orphelins

Je rappelle que le montant de l'indemnisation des SDIS, qui pallient l'absence d'autres moyens, s'élève à 123 euros par carence alors que le coût moyen qu'ils supportent est estimé entre 450 et 500 euros, tandis que ces créances sont parfois difficilement recouvrées. La proposition de loi les définit enfin. Pérenniser l'engagement des sapeurs-pompiers, c'est aussi garantir l'avenir de notre modèle de sécurité civile structuré autour du volontariat. Il s'agit donc de valoriser le volontariat. L'abaissement de cinq ans de la durée d'engagement ouvrant droit à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, l'amélioration de la prise en charge des accidents de services des sapeurs-pompiers volontaires par la sécurité sociale, la création d'un mécanisme de don de jours de congé, facilitation de l'attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » et la mise en oeuvre du mécanisme de la réduction d'impôt au titre du mécénat, au bénéfice d'un dispositif de réduction de cotisations sociales patronales, telles sont toutes les mesures que la proposition de loi porte en ce sens pour pérenniser l'engagement des sapeurs-pompiers, il faut aussi pérenniser le cadre du volontariat. Aujourd'hui, 79 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires. Nous devons faire valoir le caractère exceptionnel du volontariat dans le secteur de la sécurité civile. Non, le volontariat en matière de sécurité civile ne doit pas entrer dans le champ de la directive de 2003 sur l'aménagement du temps de travail ! Nous demanderons au Gouvernement de soumettre une réponse juridique effective à ses partenaires européens, à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Ma collègue Laurence Harribey y reviendra plus longuement dans son intervention. Pour leurs besoins d'urgence, nos concitoyens et nos concitoyennes s'adressent aux services de police et de gendarmerie, à ceux d'aide médicale urgente et aux services de sécurité civile. C'est à ce titre que la présente proposition porte l'expérimentation des plateformes « bleu-blanc-rouge », police-SAMU-pompiers. Cette expérimentation semble aller dans le sens du renforcement d'un continuum de services, mais une discussion doit avoir lieu. Nous devons aboutir à une situation qui garantisse, à la fois, aux services de sécurité civile leur pleine efficacité et aux services d'aide médicale le plein exercice de leur compétence. Le groupe Socialiste,

la proposition de loi que nous examinons est à la fois très attendue et très observée par tous les acteurs de la sécurité civile et de la santé. attendue, parce qu'elle apporte des réponses à des questions déjà anciennes et à des situations bloquées depuis trop longtemps. Elle est observée, parce qu'elle comporte des modifications significatives de l'organisation des secours, qui concernent au premier chef les personnels de terrain. La portée de ce texte n'est donc pas seulement technique. Ses véritables enjeux sont de redéfinir le service que nous voulons offrir à nos concitoyens, pour leur garantir un dispositif simple et efficace d'appel d'urgence ; la place et la reconnaissance que nous accordons à nos services de secours, à leurs victimes et au volontariat au service de l'intérêt général ; et l'équité que nous voulons garantir aux collectivités qui assument la charge financière de la carence ambulancière. En premier lieu, le texte consolide l'instauration à terme d'un dispositif d'appel d'urgence plus resserré. Cette orientation est nécessaire et positive, car- il faut le dire -ce n'est pas aux appelants de gérer la complexité à laquelle notre système d'appel est parvenu. C'est à nous de le réformer. Ce choix suscite encore un débat animé, dont la question centrale est celle de la place de la régulation médicale. Il faut savoir l'entendre, et il faudra en tenir compte dans le dispositif définitif, sans remettre en cause pour autant le principe de l'unification. Mais il faut aussi maintenant tout faire pour que des décisions soient prises. Le choix du Sénat, exprimé déjà en 2019, est de voir émerger une plateforme d'appel commune. Aujourd'hui, les rapporteurs nous proposent, à juste titre, de nous inscrire dans la logique de l'expérimentation, préconisée à l'Assemblée nationale. La commission des lois propose, en outre, de réduire de trois à deux ans le temps de cette expérimentation pour rendre plus effective l'obligation qu'elle débouche sur un dispositif nouveau. C'est une avancée importante qui marque notre volonté que l'expérimentation soit réellement conduite, qu'elle le soit avec célérité et qu'elle aboutisse. En deuxième lieu, ce texte clarifie le cadre d'intervention des services d'incendie et de secours et fait évoluer notre modèle vers une meilleure coordination avec les loi améliore la reconnaissance des pompiers, en particulier en créant une mention « Mort pour le service de la République » afin d'honorer les personnes ayant péri en accomplissant leurs missions dans des circonstances exceptionnelles. Elle reconnaît également le statut de « pupille de la République » aux enfants des défunts. C'est un juste hommage à nos 240 000 pompiers, dont 80 % sont des volontaires.

Leurs interventions sont devenues plus complexes et plus dangereuses aussi, avec la multiplication des agressions. Sans ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps au risque de leur vie, beaucoup de nos campagnes n'auraient quasiment plus de secours. Je souhaite les saluer et les remercier pour leur courage et leur engagement. En troisième lieu, le texte clarifie la définition des carences ambulancières, qui se sont multipliées et qui constituent un véritable transfert de charges de l'État vers les départements. La commission des lois est allée encore plus loin, en supprimant l'obligation de prescription médicale pour pouvoir qualifier une intervention de carence ambulancière et en clarifiant la faculté de refuser ou différer la mise en oeuvre d'une carence. Enfin, elle a introduit la possibilité de requalifier une intervention en carence ambulancière, ce qui permettra aux SDIS d'être justement indemnisés lorsqu'ils réalisent une intervention à la demande du 15 qui s'avère par la suite relever de cette catégorie. ministre, il reste désormais au Gouvernement à réitérer et à tenir son engagement de revalorisation significative du tarif national, pour rendre aux SDIS la maîtrise de leurs moyens. En conclusion, je tiens à rappeler que, dans de nombreux départements, les sapeurs-pompiers volontaires réalisent la grande majorité des interventions, soit plus de 80 % d'entre elles dans mon département de l'Indre. Il est donc juste que ce texte conforte et encourage le volontariat par des mesures incitatives pour les sapeurs-pompiers volontaires, mais également pour leurs employeurs. Cependant, l'incertitude que continue de faire peser la jurisprudence européenne sur notre régime de volontariat reste entière.

En effet, ce texte, s'il cherche à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser notamment le volontariat, est examiné dans un contexte de relative insécurité juridique

les conditions de travail de manière générale. Cependant, lorsque la Cour de justice de l'Union européenne, en application de cette directive, assimile le temps d'astreinte d'un sapeur-pompier volontaire à un temps de travail, c'est tout le modèle du volontariat

Tous soulignent la nécessité de faire évoluer la législation européenne. Les réponses sont restées embarrassées, relativement incantatoires et peu probantes. d'autant plus que la Commission européenne, où l'on ne semble pas convaincu du problème, renvoie à la possibilité pour les États d'établir des dérogations liées à la nécessité d'assurer un service continu. néanmoins- c'est une forme de « en même temps » -, dans une réponse à une question écrite, en 2018, que la notion de « travailleur » est un concept autonome de l'Union européenne, indépendant du statut en droit national. Quant à la suggestion d'une directive spécifique aux services de sécurité et de protection civile, tenant compte de la dimension volontaire et bénévole des activités, la Commission européenne répond que les dispositions actuelles du traité ne fournissent pas de base juridique pour réglementer le temps de travail des volontaires. L'« ornière », comme les rapporteurs la qualifient à juste titre, est d'autant plus corsée qu'en juillet dernier, saisie par la République slovène d'un litige entre un sous-officier et sa hiérarchie au sujet du paiement de tours de garde

l'exercice d'équilibre devient périlleux, et il existe bien un problème de définition juridique que seule une volonté politique peut déterminer. de loi Matras réaffirme et consolide le caractère volontaire citoyen, comme la notion d'engagement. Il n'empêche que la question de la sécurité juridique du modèle français de sécurité civile reste posée. Les rapporteurs ont donc sans doute raison de proposer la suppression de l'article 22 qui affirme de manière incantatoire le caractère citoyen, librement décidé et consenti de l'engagement de sapeur-pompier volontaire, et de renvoyer à la responsabilité du Gouvernement de saisir la prochaine présidence française de l'Union européenne pour avancer enfin sur cette question.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, est-il plus noble mission que d'être au service de ses concitoyens pour les protéger et sauver des vies ? Par leur action, leur sens de la solidarité et du service public, par leur goût de l'effort collectif et du dépassement de soi au service de l'intérêt général, les acteurs de la sécurité civile incarnent des valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre solidarité nationale. Mon département, le Gard, trop souvent meurtri par des événements catastrophiques, notamment les inondations et les incendies, sait ce qu'il doit à ces femmes et à ces hommes. Il sait qu'il peut compter sur eux, sur leur compétence et sur leur engagement, en toutes circonstances. C'est pour cette raison que je souhaite leur dire publiquement, ce soir, merci. Merci avec un grand « M » ! Nous oublions trop souvent de le leur dire. Mesdames, messieurs les sapeurs-pompiers, vous êtes la fierté de la France et nous vous devons respect et admiration. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la reconnaissance publique doit être à la hauteur de votre engagement. Garantir un égal accès des Français aux services d'incendie et de secours, valoriser le savoir-faire et l'expertise française en matière de sécurité civile, voilà notre mission Au quotidien, force est de constater l'efficacité de notre modèle. L'image dont jouit, à travers le monde, la sécurité civile française en témoigne. Pourtant, face à l'accroissement des sollicitations opérationnelles, à la baisse de l'engagement volontaire volontaire et à l'augmentation de l'insécurité liée aux interventions, la législation en vigueur nécessitait d'être améliorée. Cette proposition de loi s'y emploie avec justesse, et je me réjouis, à ce titre, qu'elle fasse l'objet d'un consensus aussi marqué. Cette proposition de loi porte ainsi en elle de nombreuses avancées qui viennent clarifier le cadre d'intervention des services d'incendie et de secours. Elle donne enfin une définition objective de la carence ambulancière, incite des jeunes à s'engager en rendant la formation certifiante, reconnaît le dévouement des sapeurs-pompiers en en mettant en place une mention honorifique « Mort pour le service de la République » et en créant un statut de pupille de la République, à destination des enfants de sapeurs-pompiers décédés en service commandé. Elle acte aussi l'expérimentation d'une plateforme commune de régulation des appels d'urgence. À cet égard, le choix d'une expérimentation ramenée à deux ans me paraît être une position nuancée et consensuelle qui respecte l'intérêt de tous d'aller vers une simplification. de loi comporte enfin un certain nombre de dispositions très attendues visant à mieux protéger les services de secours. Face au manque de réponse législative, certains SDIS ont dû mettre en place eux-mêmes une organisation en réponse aux menaces et outrages. Le SDIS du Gard a par exemple rédigé des outils de formation et constitué une équipe de référents formateurs exerçant auprès de leurs collègues, ainsi que des équipes de médiateurs intervenant auprès des associations qui oeuvrent dans les quartiers difficiles. Leur modèle a d'ailleurs été repris par le Centre national de la fonction publique territoriale, afin de former des sapeurs-pompiers d'autres casernes sur le territoire français. Il était temps que nos lois viennent soutenir Je souhaite appeler votre attention sur deux points, dont le premier est le volontariat. La réglementation européenne, par le biais de l'arrêt, pourrait menacer à terme notre modèle de sécurité civile, en considérant le temps d'astreinte d'un sapeur-pompier volontaire comme un temps de travail au sens de la directive européenne dite « DETT » du 4 novembre 2003. Le volontariat est pourtant au coeur du modèle de sécurité civile français. Il représente ainsi 80 % de l'ensemble des effectifs des sapeurs-pompiers, avec une très forte densité dans le milieu rural. L'application d'une telle mesure aurait ainsi de très importantes conséquences sociologiques, opérationnelles et financières. Elle serait de nature à désorganiser totalement le maillage des SDIS, à l'heure où les inégalités territoriales s'accroissent. Le volontariat, au-delà de sa vertu civique exemplaire, est l'élément central du fonctionnement du service public de sécurité civile, qui a toujours été soutenu par les parlementaires et les gouvernements depuis 2003. Nous comptons ainsi sur vous, madame la ministre, pour défendre avec vigueur le statut des sapeurs-pompiers volontaires. terminer mon propos, je veux parler du rayonnement de la France auquel notre modèle unique de sécurité civile se doit de participer. Chacun a pu constater à quel point l'entraide entre les États membres en cas de catastrophe naturelle était nécessaire. À cet égard, le projet d'installation en France, plus précisément sur la base de Nîmes-Garons, du centre d'expertise européen pour lutter contre les risques,

permettez-moi tout d'abord de m'associer aux précédents orateurs pour saluer le travail accompli par les rapporteurs de ce texte. J'ai également une pensée pour Catherine Troendlé, à qui j'ai succédé dans cet hémicycle.

Comme vous le savez, elle et moi sommes originaires du Haut-Rhin, un département qui fait figure d'exception en matière de sécurité civile puisque, dans notre pays, il est l'un des mieux pourvus en nombre de sapeurs-pompiers volontaires. À ce jour, nous comptons plus de 5 280 citoyens engagés en qualité de sapeurs-pompiers et plus de 1 300 JSP qui se destinent à prendre la relève. Nous comptons près de 190 corps de première intervention communaux et 18 CPI intercommunaux, en complément du service départemental d'incendie et de secours. Depuis la loi du 3 mai 1996 tendant à la départementalisation des services d'incendie et de secours, seuls neuf départements en France comptent encore des CPI. Pourtant, je peux témoigner que le fonctionnement conjoint des CPI et des SDIS est une richesse pour nos territoires ruraux et que les populations et les communes y sont très attachées. À ce titre, je salue l'adoption d'un amendement en commission des lois, qui vise à ouvrir à l'ensemble des conseillers municipaux la possibilité de se présenter pour devenir membre du conseil d'administration d'un

Vous l'aurez compris, dans le Haut-Rhin, la combinaison de ces deux organisations complémentaires assure un maillage de proximité qui démontre chaque jour son utilité, grâce à son efficacité et à sa rapidité d'intervention. Tous les élus de mon territoire souhaitent la pérennisation de ce modèle d'organisation qui apporte les bonnes réponses aux enjeux de sécurité civile que nous connaissons. Les CPI et les SDIS ne doivent pas s'opposer, car, ensemble, ils assurent une protection efficace de nos concitoyens face à la multiplicité des risques naturels, technologiques, sanitaires et industriels auxquels nous sommes confrontés. Pour avoir rencontré de nombreux sapeurs-pompiers de mon département ces dernières semaines, je peux attester que nous allons discuter d'un texte très attendu. Il apportera des réponses aux nouvelles missions qui leur incombent, au besoin de clarification et de meilleure articulation de leur action avec celle des services d'aide médicale d'urgence et à une attente de reconnaissance et de protection juridique pour ces hommes et ces femmes qui interviennent au quotidien, avec courage et désintéressement, en toutes circonstances, et parfois au péril de leur vie. la valorisation du volontariat est un enjeu essentiel qui mérite d'être amélioré, en permettant par exemple une reconnaissance de cette formation au même titre que d'autres enseignements facultatifs. C'est pourquoi je vous proposerai un amendement afin que les JSP puissent obtenir des points bonus pour le brevet des collèges et le baccalauréat, lorsqu'ils ont validé leur formation de sapeurs-pompiers volontaires. J'espère vraiment que vous le voterez. La seule ombre au tableau reste le risque de déstabilisation juridique qui pèse sur notre modèle de secours, du fait de la directive européenne sur le temps de travail. Je crois savoir que le Gouvernement a reçu des gages de l'Union européenne pour que les sapeurs-pompiers volontaires n'y soient pas soumis. J'espère, madame la ministre, que vous pourrez nous le confirmer. La discussion

Si cet article est adopté, les services d'incendie et de secours auront une mission supplémentaire à assumer. En plus des secours dont ils ont en toute logique la charge,

Le présent amendement tend à supprimer l'article 2 au motif que celui-ci ouvre la possibilité aux sapeurs-pompiers d'accomplir certains soins d'urgence. Nous sommes défavorables à la suppression de cet article pour deux raisons. La première est qu'il permet d'expliciter les missions des services d'incendie et de secours et que c'est sur la base de cette définition que l'article 3 de la proposition de loi permet aux SDIS de différer ou de refuser une intervention qui ne relève pas de leurs compétences. Les pompiers ne sont pas les factotums des autres services publics, et il est temps que la loi le reconnaisse. La seconde raison est que la pratique de certains soins d'urgence, limitativement énumérés par décret,

Guidez. L'alinéa 3 de cet article, inséré par les députés, prévoit que les sapeurs-pompiers peuvent participer à la mise en place d'activités de télémédecine dans le cadre de leurs compétences. La télémédecine, dont le covid-19 a permis un développement très récent, consiste en un ensemble d'actes qui nécessite une lecture et une analyse de données de santé par un professionnel de santé ayant suivi trois années d'études. Ce terme reste donc beaucoup trop générique et laisse entrevoir la possibilité de réaliser des actes relevant de professions réglementées.

Benarroche, sur l'article. Je souhaite profiter de cet article, qui actualise les références applicables aux brigades militaires de Paris et de Marseille, pour évoquer l'enjeu important de la sécurité dans les ports. ports. Chacun connaît l'évolution significative de l'activité des ports depuis quelques années, que ce soit dans le transport de porte-conteneurs ou dans le développement exponentiel de l'activité de croisière. ces sites accueillent tout type de marchandises sensibles- hydrocarbures, vrac liquide, vrac solide, etc. -et abritent de plus en plus différents types d'industries : raffineries, sidérurgies ou industries chimiques.

Aussi, malgré la faible occurrence à ce jour des incidents de ce type- heureusement ! -, la lutte contre ces sinistres exige des moyens spécifiques au milieu portuaire. Aujourd'hui, seule une circulaire datant de 1977, cosignée par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, donne des orientations en matière de prévention et de lutte contre les incendies dans les ports. ne prend toutefois en compte les évolutions de l'organisation des SDIS ni les apports successifs de plusieurs textes, dont le décret Orsec issu de la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004. En outre, sa force probatoire fait débat, car elle n'a pas été publiée.

qui s'étend sur plusieurs villes, rien ne permet de déterminer quelles sont les responsabilités des différentes communes. Le travail en question pointait la nécessité d'une évaluation des besoins et des moyens pour ces risques spécifiques. À l'occasion de l'examen de cette proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile, je souhaite vous alerter, madame la ministre, sur les difficultés qu'ont les forces de sécurité, en particulier les marins-pompiers, par exemple dans le port de Marseille, à affronter ces nouveaux risques de plus en plus importants, importants, en raison d'un manque de réflexion globale sur l'organisation de la sécurité dans les ports. Je demande donc au Gouvernement d'inscrire à son agenda une étude sur la sécurité dans les ports et la façon d'assurer la sécurité civile dans ces zones portuaires.

de Marseille et son amiral, d'apporter des corrections de coordination prenant en compte la spécificité des missions qui sont les siennes. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille a comme responsabilité la sécurité sur la ville de Marseille, sur le grand port maritime de Marseille et sur le parc naturel des Calanques.

amendement vise à expliciter la compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans les emprises des aéroports parisiens, y compris pour les parties de ces emprises situées en grande couronne.

de temporiser le départ en mission et, éventuellement, de requalifier une intervention dont la carence n'aurait pas été identifiée au départ. L'article 3 permet d'y répondre. Le second enjeu est celui de l'organisation globale du transport sanitaire. Or une réforme du transport sanitaire urgent est en cours, certes avec une sollicitation tardive des élus locaux. Elle pourrait conduire à la suppression des gardes ambulancières dans certains départements. Dans l'attente d'un travail en commun avec les ministères de l'intérieur et de la santé, l'Assemblée des départements de France s'oppose vivement à une désertification des territoires, en particulier les plus ruraux, en termes de garde ambulancière. La problématique soulevée par les transports sanitaires dans le cadre des secours à la personne est réelle. Il arrive que la coordination entre les différents opérateurs se fasse en bonne intelligence, permettant ainsi d'éviter les écueils d'une opérationnalité moindre pour les SIS, quand trop de leurs équipements sont sollicités pour de telles tâches. Il nous apparaît donc essentiel de rappeler la nécessaire coordination des différents opérateurs, en insistant sur la part que doivent prendre les services d'ambulances privées, notamment dans le cadre de garde ambulancière. Les SIS ne peuvent être considérés comme les opérateurs uniques des soins d'urgence et doivent ainsi se coordonner avec les autres acteurs comme le SAMU et les SMUR. L'intervention des SDIS pour répondre à des carences ambulancières ne saurait conduire, pour autant, à la suppression des gardes ambulancières dans certains départements. ? Ces deux amendements sont similaires et visent à préciser dans la loi que, dans l'organisation de l'aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire, les services d'incendie et de secours ne sauraient être considérés comme des opérateurs uniques. Ils tendent également que les SDIS ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières. Nous sommes d'accord sur le principe : les SDIS ne sauraient être considérés comme les opérateurs uniques des soins d'urgence, et le transport sanitaire ne correspond pas à leur coeur de métier. On ne peut que regretter que l'organisation du transport sanitaire repose parfois sur les services d'incendie et de secours et la réalisation de carences ambulancières. Sur le plan juridique toutefois, le dispositif proposé ne me paraît pas opérationnel. L'article 3 de la proposition de loi précise déjà que les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux opérations de secours se rattachant directement à leurs missions de service public. Il produit donc les mêmes effets. La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

commission ? Cet amendement ne rejoint sur aucun point la position de la commission. L'avis est donc défavorable. La possibilité de requalification des carences ambulancières est absolument incontournable. Elle permet aux SDIS d'être justement indemnisés lorsqu'ils ont réalisé une intervention à la demande du 15 dont il est avéré qu'elle relevait en pratique de la carence. Cela permet de répondre aux imperfections d'un système où l'appréciation de la carence relève principalement du médecin régulateur du SAMU et où l'indemnisation des sapeurs-pompiers est très en deçà du coût réel- 124 euros,

à Mme Jocelyne Guidez. Il est proposé que l'association départementale des transports sanitaires urgents soit consultée par le service d'aide médicale urgente pour constater le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés. La rédaction de l'Assemblée nationale est contraire à l'avenant n° 10 de la réforme de la tarification de l'assurance maladie. Il est impossible de laisser les pompiers seuls avec le SAMU valider les carences, même après la réalisation de l'intervention, comme prévu à l'alinéa 7 de la proposition de loi.

Mes chers collègues, les services d'incendie et de secours, hélas ! comme beaucoup de nos compatriotes qui portent un uniforme, sont le plus souvent la cible d'attaques injustifiées. Dans cette période éprouvante, nous devons plus que jamais les soutenir. L'adoption de cet amendement serait une façon concrète de le faire. est l'avis de la commission ? Mme Bonfanti-Dossat propose que les sapeurs-pompiers puissent utiliser gratuitement le réseau routier et autoroutier en intervention. Nous sommes complètement d'accord, mais cela est déjà prévu par le code de la voirie routière. Son article L. 122-4-3 dispose explicitement que « les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération ne sont pas assujettis au péage ». L'article 3 ne fait que préciser les modalités de mise en oeuvre de ce principe. S'agissant de l'exonération des amendes en cas d'excès de vitesse capté par des radars fixes en intervention, cela ne me paraît pas opportun. Dans la pratique, les véhicules d'urgence sont flashés comme tout usager, et les services peuvent demander l'annulation de l'amende en justifiant du caractère opérationnel de l'intervention. Ce système est équilibré. Il permet de concilier l'égalité des usagers devant la loi et la nécessité de prévoir des dérogations pour les véhicules d'urgence.

Cet amendement vise à supprimer le IV de l'article 3, puisqu'il est impossible de contrôler les prestations réalisées au bénéfice des SMUR s'il n'y a pas de centralisation des prestations auprès du siège de l'hôpital détenteur du service d'aide médicale urgente. Aujourd'hui, cette centralisation des prestations n'existant pas, l'adoption d'une telle disposition ne reviendrait qu'à codifier une disposition totalement inapplicable dans les faits. Je vous rejoins sur le fait que la prise en charge par les établissements de santé des moyens engagés par les SDIS au profit des SMUR peut être complexe à mettre en place selon l'organisation des services sur le terrain. Néanmoins, cela ne justifie pas de faire peser cette charge sur les SDIS, alors que ce sont eux qui mettent à disposition leurs moyens. Ensuite, il me semble que c'est tout l'intérêt du système conventionnel prévu par cet article. Il offre une souplesse suffisante aux acteurs locaux pour s'adapter à l'organisation locale des SMUR et permettre une répartition équitable de la charge. La commission demande le retrait de cet amendement

Le présent amendement vise à étendre l'applicabilité des mesures législatives prévues pour les services départementaux d'incendie et de secours aux services territoriaux d'incendie et de secours. Il vise également à prévoir une mesure d'ordre rédactionnel. Quel est l'avis du Gouvernement ? Favorable.

stratégique de l'État et la hiérarchie financière et technique du département. J'ajoute que les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires publics territoriaux. Au-delà des

mais je rappelle que la création de ce système ...

Le présent amendement tend à supprimer l'article 5 de la proposition de loi, qui permet, avec l'article 4, de rationaliser en trois catégories les différents services d'incendie et de secours.

L'information préventive de nos concitoyens constitue le premier maillon de la résilience d'une population. La connaissance des risques auxquels elle peut se trouver confrontée est fondamentale- je l'évoquais dans mon intervention en

Quel est l'avis de la commission ? Le présent amendement tend à ce que les communes concernées par un risque majeur contribuent à l'information de leur population quant au risque majeur qui les menace. Il offre un cadre légal et assure des garanties minimales pour les populations concernées. Certaines zones sont soumises à des risques clairement identifiés, et l'apprentissage des bons réflexes par la population peut clairement contribuer à sauver des vies. La commission a donc émis un avis favorable.

: La parole est à M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités de suivi du plan communal de sauvegarde et à assurer la coordination avec la nouvelle fonction de correspondant incendie et secours prévue par l'article 8 A de la proposition de loi. Il précise que le suivi du plan peut être assuré par un adjoint ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile et désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours. Cela est cohérent avec l'amendement n° 154 que nous présenterons à l'article 8 A et qui vise à prévoir la création d'un correspondant incendie et secours dans le seul cas où aucun adjoint ou conseiller municipal n'a été chargé des questions de sécurité civile en application de l'article L. 731-1 du code de la sécurité intérieure.

Les retours d'expérience ont montré l'utilité et l'efficacité de ces dispositifs, qui apportent une réponse locale, au plus près des populations et de la réalité du territoire.

Nous vous proposons d'étendre l'obligation de réalisation d'un PCS à d'autres risques, dont l'intensité ou la soudaineté rend nécessaire l'existence d'un tel plan, en ce qu'il permet la mise en place rapide de mesures de sauvegarde et de protection des populations.

commission ? Le présent amendement tend à étendre les catégories de risques rendant obligatoire un plan communal de sauvegarde. Nous pensons que cette extension est la bienvenue, car les risques naturels ne sont pas les seuls à devoir être pris en compte à l'échelle communale ou intercommunale pour apporter un meilleur appui aux populations. En outre, les plans communaux de sauvegarde existants ont montré leur efficacité pour organiser la réaction à des sinistres d'ampleur, et cette efficacité sera encore accrue par la mise en place d'exercices réguliers prévue par l'article 6 de ce texte. L'avis est donc favorable.

Mme Maryse Carrère. L'article 6 de cette proposition de loi rend obligatoire l'adoption d'un plan intercommunal de sauvegarde pour les EPCI à fiscalité propre, dès lors qu'au moins une des communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde. Nous comprenons le sens de cette disposition, mais une telle obligation nous paraît excessivement contraignante pour l'intercommunalité, d'autant que la

L'article 6 rend ce plan obligatoire, dès lors qu'une commune de l'EPCI est dans l'obligation de se doter, elle-même, d'un plan de sauvegarde. Nous soutenons le dispositif de l'article 6, car les plans de sauvegarde doivent notamment prévoir les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes et la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Or un sinistre d'ampleur prévu dans un PPRN qui toucherait une commune aurait également un impact sur les communes voisines, et il est important que ces réponses soient effectives à l'échelle de l'EPCI auquel elle appartient. C'est pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

coordination. L'amendement n° 18 rectifié est contraire à la position de la commission. Il vise à modifier la rédaction de l'article 8, qui complète le code de la sécurité intérieure afin de préciser les cas exorbitants dans lesquels le préfet se substitue au maire pour assurer la direction des opérations de secours. Il vient notamment supprimer le pouvoir de réquisition des préfets en cas de crise majeure au profit d'une faculté de simple association des personnes et de leurs moyens. Or nous savons que les préfets n'utilisent ce pouvoir qu'en cas d'extrême nécessité. Les en priver pourrait se révéler dangereux en cas de crise sévère.

Cet amendement vise à rappeler que la gestion des situations de crise relève aussi bien du représentant de l'État que du maire. La précision que nous proposons d'insérer au sein de l'article 8 de la proposition de loi nous paraît utile à plus d'un titre. Cet article crée un nouveau cadre juridique dans lequel la direction des opérations serait directement confiée au représentant de l'État dans le département en cas de crise exceptionnelle. Cependant, la notion de crise exceptionnelle n'est pas précisée. Ce choix rédactionnel laisse penser que l'on s'oriente vers une extension du champ d'intervention du préfet, qui serait susceptible d'agir pour différentes catégories de crise, au-delà des crises de sécurité civile. Dans un texte relatif à la sécurité civile, il aurait été préférable d'éviter le mélange des genres avec les crises de sécurité publique, qui reposent sur d'autres ressorts et l'intervention d'autres acteurs. La lisibilité de l'action publique aurait mérité davantage de rigueur à cet égard.

se fait « sans préjudice des pouvoirs du maire dans la gestion des opérations de secours ».

M. le rapporteur. Le présent amendement vise à préciser les conditions de création d'un correspondant incendie et secours au sein du conseil municipal. Afin d'éviter toute redondance, il tend à préciser qu'un tel correspondant n'est désigné que dans l'hypothèse où n'a pas déjà désigné un adjoint ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. En cohérence avec l'article 2 de la proposition de loi, cet amendement a également pour objet d'étendre les missions d'information et de sensibilisation du correspondant aux soins d'urgence. Enfin, il vise à procéder à une coordination.

rectifié. En concertation avec les rapporteurs, je propose une rédaction plus opérationnelle en ce qui concerne la composition du bureau et du conseil d'administration des SDIS, en redéfinissant les conditions d'élection à la fonction de vice-président. Puisque nous choisissons de ne pas restreindre l'élection au conseil d'administration aux seuls maires et maires adjoints, il est logique d'autoriser adjoints, il est logique d'autoriser les conseillers municipaux à intégrer le bureau du conseil d'administration du SDIS. Actuellement, une place de vice-président sur les existantes est réservée de droit au collège des maires. L'amendement vise à élargir cette priorité à l'ensemble des représentants des communes, ce qui garantirait une meilleure représentation des communes et des EPCI au sein du conseil d'administration des SDIS, quand bien même aucun maire n'y serait élu.

vise à tirer les conséquences du nouvel article 8 B introduit en commission, qui permet à tous les conseillers municipaux de se présenter à l'élection au conseil d'administration du SDIS. du SDIS. Il procède de la même logique pour l'élection au bureau du conseil d'administration. Actuellement, une place de vice-président sur les trois existantes est réservée de droit au collège des maires. Il s'agit de transférer cette priorité des seuls maires vers l'ensemble des représentants des communes et des EPCI. donne ainsi davantage de libertés aux conseils d'administration des SDIS pour s'organiser et il leur permet de valoriser au mieux l'expertise disponible. En effet, de nombreux conseillers municipaux et communautaires disposent d'une expertise très poussée en matière d'incendie et de secours. Il est donc logique et légitime que cette priorité

Année après année, nous observons que le nombre de feux de forêt augmente et que les incendies se répandent dans des régions jusque-là épargnées. Les forêts du sud de la France ne sont plus les seules concernées. Il est donc indispensable qu'un diagnostic du risque soit désormais inclus dans les SDACR afin que les moyens de lutte mis en oeuvre sur le terrain soient adaptés.

d'un dispositif d'alerte des populations les opérateurs de téléphonie. Toutefois, les travaux de transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ont abouti au cours de la navette parlementaire. Ainsi a été publiée l'ordonnance du 26 mai 2021, qui consacre ce dispositif. Le Gouvernement propose aujourd'hui au Sénat de procéder à la ratification de l'article 3 de cette ordonnance. Ce vote permettra de souligner l'action résolue de la France pour concrétiser le projet de système

Ce sous-amendement vise à préciser que la ratification proposée ne porte que sur le de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021

Orange, des carences du dispositif d'acheminement des appels d'urgence ont été mises en exergue, notamment l'absence de supervision spécifique pour les numéros d'urgence. Le rapport d'évaluation réalisé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) le 19 juillet 2021 a souligné la nécessité de réformer, pour mieux le sécuriser, le cadre légal relatif à l'acheminement des appels d'urgence. Le présent amendement constitue une réponse aux recommandations de ce rapport. Il vise à renforcer, en la clarifiant, l'obligation d'acheminement des communications d'urgence figurant au du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Il vise également à compléter cette obligation, en imposant la mise en place d'une supervision technique des dispositifs de communication d'urgence permettant une remontée d'alerte dans de meilleurs délais. Quel ? Cet amendement a pour objet de répondre à la panne des numéros d'urgence survenue au mois de juin dernier. Il tend à approfondir les obligations qui pèsent sur les opérateurs afin qu'ils mettent en oeuvre toutes mesures permettant de garantir

accéder aux informations du SIV. Le développement des outils numériques de terrain est tel que l'utilisation de ces informations, directement sur le terrain, j'y insiste, sera de nature à faciliter l'intervention en sécurité des forces de sécurité civile. Le second pour garantir l'accès à ce même système des personnels de l'Agence du numérique de la sécurité civile, en charge du développement et de la maintenance de ces outils à destination des SDIS. Il est indispensable de pouvoir vérifier la parfaite intégration technique des connecteurs dans les outils opérationnels. Il reste bien évidemment entendu que ces accès, tant des sapeurs-pompiers que des équipes techniques, resteront soumis aux très fortes contraintes de sécurité liées à l'accès au SIV. Le sous-amendement

les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers pourraient consulter le SIV lorsqu'ils exercent des missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur. le Gouvernement vise les personnels habilités du prestataire autorisé par l'État, en charge du développement, de la maintenance et de l'exploitation des systèmes et applications nécessaires à l'exercice de ces missions. Sur la première catégorie, les pompiers, il nous apparaît légitime que ceux-ci puissent savoir à qui appartient un véhicule dans le cadre de leur mission de sécurité civile. Toutefois, les contours des missions de sécurité civile pour lesquelles cet accès est mis en place devraient être précisés, de même que les données auxquelles les pompiers ont accès. La seconde catégorie est, elle, beaucoup plus problématique. En effet, ni le texte ni l'objet de l'amendement n'expliquent en quoi un tel accès serait utile. Un prestataire chargé du développement et de la maintenance n'a, en principe, pas besoin d'accéder au traitement des données à proprement parler pour réaliser ses missions. De plus, cette référence est imprécise et recouvre potentiellement un grand nombre de personnes. Nous présentons donc un sous-amendement visant à retirer

reprendre, puissent accéder aux données pour garantir le développement et la maintenance des connecteurs avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV). L'augmentation du niveau de sécurité offert par l'accès aux données va permettre de mieux protéger les sapeurs-pompiers des accidents

pour tester régulièrement le bon fonctionnement de l'outil. L'habilitation mentionnée ne sera délivrée par le directeur de l'ANSC qu'à un nombre très restreint de personnels, limitant ainsi au strict nécessaire l'accès aux données. Les outils de développement informatique utilisés par l'Agence nécessitent une identification, un nom d'utilisateur et un mot de passe spécial pour accéder au réseau, afin de suivre l'activité des agents en cas de besoin. Je voudrais aussi préciser ici que ces agents sont, par ailleurs, soumis au respect des règles de traitement des données personnelles, conformément au règlement général sur la protection des données. Pour rappel, l'article L. 330-2 du code de la route autorise, par exemple, l'accès aux données du SIV des agents chargés du traitement des appels d'urgence, à seule fin d'identifier un véhicule, et ce conformément aux dispositions du Règlement délégué n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012, qui complète les directives du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne notamment la mise à disposition harmonisée d'un service d'appels d'urgence au bénéfice d'agents de droit privé travaillant dans des plateformes de téléassistance. Aussi, nous vous proposons, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre sous-amendement, faute de quoi je serai contrainte d'y donner un avis défavorable.

lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, autorise de manière permanente les personnels des forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, et des services d'incendie et de secours à accéder aux parties communes d'immeubles lors de leurs interventions. Avec cette disposition, les propriétaires ou les exploitants devraient assurer un tel accès. Actuellement, la police et la gendarmerie peuvent être autorisées

pour les forces de sécurité intérieure et les pompiers. Alors que nous examinons un texte portant sur les services d'incendie et de secours, nous préférons circonscrire cette obligation d'accès obligation d'accès aux seuls pompiers. Au regard des missions qu'ils réalisent, qui sont différentes de celles des forces de sécurité intérieure, cet accès nous semble bien justifié pour les services d'incendie et de secours. Cependant, nous ne souhaitons pas que ce dispositif soit étendu aux forces de sécurité intérieure, sachant que les parties communes demeurent- faut-il le rappeler ? -un lieu privé. Pour résumer, nous proposons de limiter aux seuls pompiers la possibilité d'accéder aux parties communes d'immeubles sans autorisation préalable et de maintenir le régime actuel pour les forces de sécurité intérieure, qui bénéficient déjà de dérogations juridiques possibles.

nouvelle rédaction mêle dans un même dispositif des mesures de sécurité civile et des mesures de sécurité intérieure, ce qui est totalement différent. Il nous semble que les conséquences en matière de responsabilité n'ont pas été mesurées en cas de défaut d'application de la pour quelque cause que ce soit. En effet, il est proposé de remplacer le principe de l'autorisation d'accès par une obligation d'assurer l'effectivité de cet accès, à la charge des propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation, sans prévoir de sanction en cas de défaut de mise en oeuvre. Qu'en est-il du régime de responsabilité applicable dans ce cas d'espèce ? Le texte ne le dit pas. Par ailleurs, il est établi par une jurisprudence constante que les parties communes d'un immeuble sont des lieux privés qui ne sont ouverts à personne, sauf autorisation de ceux qui les occupent de manière permanente ou temporaire. Il nous semble préférable d'en rester au droit en vigueur, qui prévoit que les forces de police, de gendarmerie et, le cas échéant, la police municipale ont la possibilité d'intervenir de façon permanente dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation à la condition d'y avoir été autorisées par les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants. Il faut également savoir qu'en matière de police judiciaire, en particulier en cas d'enquête de flagrance, les forces de sécurité intérieure ont le droit de prendre toute mesure appropriée et pourront pénétrer dans les parties communes sans avoir besoin d'une autorisation préalable. Ne mêlons pas missions de sécurité intérieure et missions

les forces de sécurité intérieure, tout comme les pompiers, à accéder aux parties communes des immeubles à des fins d'intervention. Nos collègues proposent de s'en tenir au droit existant pour les policiers et les gendarmes et de maintenir le principe d'une autorisation par le par le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble. Cette autorisation doit toutefois être régulièrement renouvelée, alors qu'elle est, de manière générale, systématiquement accordée. Une simplification de la procédure est donc apparue pertinente à la commission. C'est pourquoi son avis est défavorable sur ces deux amendements.

est à Mme Laurence Harribey. Avec cet amendement, nous proposons une solution d'aménagement des SDIS pour les communes rurales, en permettant l'institution de centres de secours constitués de plusieurs casernes existantes. Dans certains territoires, nous le savons tous, il peut y avoir des casernes de petite taille relativement anciennes et difficiles à rénover. Plutôt que de procéder systématiquement à un regroupement complexe à mettre en oeuvre et qui passe parfois par la construction coûteuse d'un centre d'incendie et de secours, il serait plus rationnel d'ouvrir la possibilité d'instituer le principe d'un centre de secours constitué de plusieurs casernes existantes. C'est une forme de mutualisation. mutualisation. Cette mesure serait de nature à garantir le maintien de casernes de proximité, mais nous souhaitons aussi nous inscrire dans la définition essentiellement opérationnelle du centre d'incendie et de secours, au sens des dispositions qui régissent le service public d'incendie et de secours. Quel

Comme vous le savez, l'article 12 de la proposition de loi entend supprimer la nomenclature distinguant centres de secours principaux, centres de secours et centres de premiers secours. Cette simplification est la bienvenue. Or cet amendement semble aller à l'encontre de cette logique. De surcroît,

Nous proposons ainsi d'intégrer de manière explicite au sein de l'article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales les personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein du corps départemental au sein du corps départemental des services d'incendie, tout en conservant l'ajout effectué par la proposition de loi sur le volontariat en service civique des sapeurs-pompiers. Cet article définit la composition du corps départemental des sapeurs-pompiers, avec des sapeurs-pompiers professionnels, des volontaires et des auxiliaires. Nous reprenons cet amendement, que nous avions déposé une première fois en commission et qui avait été rejeté au motif que les PATS n'ont pas vocation à rester de façon permanente et définitive au sein du SDIS dans lequel ils ont été affectés, contrairement aux sapeurs-pompiers professionnels. Il est vrai que les PATS appartiennent à des filières administratives, techniques et à des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale propres, dotés de statuts particuliers, de grilles indiciaires et de régimes indemnitaires distincts de ceux des sapeurs-pompiers professionnels. Selon nous, cette différence statutaire ne constitue pas un critère rédhibitoire justifiant de les écarter. Les PATS ne se retrouvent pas là par hasard, au gré d'une mutation ou d'un changement de poste. Ils ont accompli une démarche volontaire en candidatant à l'emploi vacant au sein du SDIS. Les contractuels ont agi de la même façon, dans le même esprit d'intégration. Au quotidien, il existe bien un esprit de corps, car ces personnels partagent les valeurs des sapeurs-pompiers et travaillent quotidiennement auprès d'eux afin d'assurer le bon exercice de leur mission. En outre, cette mesure s'inscrit en cohérence avec l'article 18 de la proposition de loi, qui ouvre la possibilité aux membres des PATS d'accéder aux emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours et qui prévoit qu'ils seront nommés conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil administration du SDIS. Sur ce dernier point, nos rapporteurs n'ont pas exprimé d'opposition à l'inscription dans le code général des collectivités territoriales des dispositions spécifiques aux membres des PATS. Nous estimons que cette intégration serait, au contraire, fort opportune. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'adopter cet amendement. L'amendement de mon collègue, cet amendement vise à intégrer les personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein du corps départemental de sapeurs-pompiers. Il s'agit en effet de personnels absolument essentiels au bon fonctionnement des services. Cette intégration, outre qu'elle interviendrait comme une clarification juridique et administrative très attendue de leur situation, serait aussi la reconnaissance symbolique de l'appartenance commune de ces femmes et de ces hommes au corps des sapeurs-pompiers. Si cet amendement ne devait pas être adopté, il serait souhaitable de pousser la réflexion sur les conditions de l'abolition de la distinction surannée entre opérationnels et administratifs.

des effectifs. Le Sénat lui-même a d'ailleurs oeuvré pour le renforcement de leur intégration au fonctionnement des SDIS. La proposition de loi déposée par Mme Catherine Troendlé et adoptée en 2019 avait permis aux membres des PATS de désigner un représentant

D'après son objet, cet amendement vise à revenir sur la création d'emplois fonctionnels de sous-directeurs au sein des SDIS. Or l'article 12 , tel qu'il a été adopté par la commission, prévoit, certes,

une fonction reconnue par les SDIS. En effet, elle va priver nos collectivités locales et nos SDIS d'une expertise précieuse. C'est d'autant plus paradoxal qu'on leur demande d'être responsables financièrement, de surveiller leurs comptes, alors qu'on les ampute d'un appui capital. Nous avons besoin de maintenir tout ce qui contribue à l'efficacité de ces services et non de supprimer une fonction nécessaire à leur logistique quotidienne. Les directeurs administratifs et financiers ne doivent donc pas être supprimés, sous peine de fragiliser le fonctionnement des services départementaux d'incendie et

Si la sous-direction Santé est la seule sous-direction explicitement prévue par la loi, il n'en restera pas moins possible de mettre en place une sous-direction chargée des affaires administratives et financières. Dès lors, le rôle important qu'assure actuellement le directeur administratif et financier

Quel est l'avis du Gouvernement ? Je voudrais préciser que les articles 12 et 12 de la proposition de loi ajustent l'organisation interne des services d'incendie et de secours, avec une organisation qui repose sur l'architecture suivante : des services de centres d'incendie et de secours, qui peuvent être regroupés au sein de groupements, eux-mêmes regroupés en sous-directions. L'article 12 vient apporter une nécessaire clarification et, surtout, un schéma d'architecture partagé, avec la création de ces sous-directions, qui amène nécessairement à la création des emplois de sous-directeur et à la prise en compte dans la chaîne hiérarchique des SIS et des délégataires. Cette disposition ne remet pas du tout en cause l'implication des responsables administratifs et financiers, qu'ils soient sapeurs-pompiers ou personnels administratifs, dès lors qu'ils sont présents dans l'organisation du SIS. Les services d'incendie et de secours peuvent tout à fait prévoir la création d'un sous-directeur administratif et financier, en cohérence avec la nouvelle structure ainsi définie. Nous sommes donc défavorables

Mme Toine Bourrat. Le présent amendement vise à ce que la composition de l'Agence régionale de santé intègre l'ensemble des acteurs du soin, parmi lesquels les sapeurs-pompiers volontaires, et qu'elle reflète ainsi la réalité de l'organisation de la politique de santé sur le territoire. Alors que le secours à la personne s'impose aujourd'hui comme le motif de sortie de secours le plus fréquent pour les SDIS, il apparaît indispensable de faire évoluer la loi pour tenir compte de cette mutation. Il s'agit ainsi d'assurer la représentation du président du conseil d'administration du SDIS au sein du conseil de surveillance de l'ARS, ce dernier ayant pour but d'émettre un avis sur le projet régional de santé, auquel les sapeurs-pompiers sont associés. est l'avis de la commission ? Le présent amendement tend à ce que les présidents des conseils de surveillance des SDIS soient représentés au sein des conseils de surveillance des ARS. Nous sommes tout à fait d'accord avec la nécessité d'améliorer la communication entre les ARS et les présidents de SDIS et saluons l'esprit constructif de cet amendement. Néanmoins, son adoption conduirait à inclure un grand nombre de nouveaux membres au sein des conseils de surveillance des ARS, c'est-à-dire autant que de départements et de SDIS dans la région concernée : 13 en Auvergne-Rhône-Alpes et 12 en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine, par exemple. C'est pour cette raison que nous demandons le retrait de l'amendement, faute de quoi nous émettrons un avis défavorable.

Cette instance peut transmettre des recommandations sur la mise en oeuvre et l'évolution de la politique de santé dans la région et sur les territoires. Le maillage dont disposent les SDIS les rend tout à fait légitimes pour siéger au sein de cet organisme, et ce d'autant plus que l'évolution de leurs missions les conduit à pratiquer principalement du secours à la personne.